la demande du groupe de l'UDI-UC, la discussion de la proposition de loi visant à assurer la sincérité et la fiabilité des comptes des collectivités territoriales, présentée par M. Vincent Delahaye

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je constate que cette proposition de loi a déplacé les foules

visant à assurer la sincérité et la fiabilité des comptes des collectivités territoriales. Aux termes de l'article 47-2 de la Constitution, « Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. En pratique, il n'est pas aisé de répondre à cette exigence légitime et la fiabilité des comptes locaux reste perfectible, malgré l'implication constante des élus, des agents territoriaux, des comptables publics et des chambres régionales et territoriales des comptes.

Ces dispositions concerneraient environ 150 collectivités territoriales et établissements publics, disposant de recettes annuelles supérieures à 200 millions d'euros, et près de 400 collectivités territoriales ou établissements, disposant de recettes annuelles comprises entre 100 millions d'euros Le texte prévoit, en outre, une saisine automatique du ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière lorsque les CRC constatent, à l'occasion d'un contrôle de gestion ou d'un contrôle de l'annualité budgétaire, une des infractions sanctionnées par cette juridiction. de loi tend ainsi à élargir les possibilités de sanction des élus locaux devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Le droit applicable aux élus locaux serait aligné sur celui qui concerne les membres des cabinets ministériels ou les administrateurs des entreprises publiques. Les membres du Gouvernement, les administrateurs élus des organismes de protection sociale et les administrateurs et agents des associations de bienfaisance resteraient hors du champ de compétence de cette juridiction. l'article 1 vise également à supprimer le dispositif de l'« ordre écrit » pour les fonctionnaires ou agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Ce mécanisme resterait toutefois applicable aux membres des cabinets ministériels, aux fonctionnaires ou agents civils ou militaires de l'État, ainsi qu'aux représentants des organismes soumis au contrôle des juridictions financières. L'article 2 de la proposition de loi prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes détentrices d'un mandat exécutif local peuvent s'assurer contre le risque de sanctions pécuniaires, sans toutefois préciser le mécanisme retenu. La Cour de discipline budgétaire et financière pourrait également prononcer une peine d'inéligibilité contre les élus locaux ayant commis une des infractions prévues par le code des juridictions financières. Il s'agirait là d'un quatrième type d'inéligibilité. Cette disposition modifierait substantiellement l'office de cette juridiction qui ne prononce, en l'état du droit, que des sanctions pécuniaires.

Les questions soulevées par ce texte ne sont pas dénuées d'intérêt et il est sans doute nécessaire de poursuivre les efforts de fiabilisation des comptes locaux. Depuis les années 1980, les règles budgétaires et comptables des collectivités territoriales ont été progressivement et utilement renforcées. Les procédures sont bien encadrées et divers contrôles sont exercés. Ainsi, le comptable public réalise des contrôles internes. Il procède à des « contrôles comptables automatisés » et transmet à l'ordonnateur un « indice de qualité des comptes locaux Les documents budgétaires et comptables sont, dès leur adoption, transmis au préfet du département qui peut lui aussi procéder à un contrôle budgétaire. Les CRC exercent deux contrôles non juridictionnels, les contrôles budgétaires et les contrôles de gestion, qui peuvent les conduire à saisir le procureur de la République, le procureur général près la Cour des comptes et aussi le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Par ailleurs, un comité national relatif à la fiabilité des comptes publics locaux a été installé en 2010. Présidé par le directeur général des finances publiques, il élabore des guides pratiques consultables en ligne. En 2014, le Gouvernement, les présidents des associations d'élus et la Cour des comptes ont signé la charte nationale relative à la fiabilité des comptes locaux pour donner plus de visibilité aux travaux de ce comité. Plus récemment, la loi NOTRe a renforcé les obligations budgétaires et comptables. Ainsi, son article 107 prévoit, par exemple, la présentation d'une étude d'impact financière pour « toute opération exceptionnelle d'investissement et, pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants, la rédaction d'un rapport annuel sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés et la structure de la dette. loi vise aussi à généraliser d'ici au mois d'août 2019 l'envoi dématérialisé des documents adressés au comptable public par les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants.

Enfin, une expérimentation est également prévue par l'article 110 de cette même loi. Elle sera conduite entre 2017 et 2023 par la Cour des comptes, en lien avec les chambres régionales des comptes, et concernera 25 collectivités volontaires. Il s'agit d'expérimenter des « dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes » et d'établir « les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local Les travaux commenceront en 2017. Un premier exercice de certification est prévu en 2020. Le Gouvernement établira un bilan d'étape en 2018, puis un bilan final en 2023. Dans son rapport annuel sur les finances publiques locales de 2015, la Cour des comptes souligne que la fiabilité des comptes du secteur local reste « imparfaite ». Elle mentionne, à l'instar des auteurs de la proposition de loi, « le défaut ou l'insuffisance de rattachement des charges et des produits [ ...] fréquemment constaté par les chambres régionales D'autres difficultés sont aussi soulevées par la Cour des comptes : un amortissement insuffisant des immobilisations, des provisions pour risques et charges trop faibles, des informations lacunaires sur la structure de la dette, etc. Dans ce contexte, nous pouvons nous interroger sur l'articulation entre le contrôle de l'annualité budgétaire qui serait créé par l'adoption de la et l'expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales. À ce stade, il semble préférable d'attendre le bilan d'étape de l'expérimentation de certification des comptes, dont la publication est prévue en 2018, ailleurs, nous nous sommes posé des questions sur les moyens à mettre en oeuvre. Est-il opportun de fixer un programme de contrôle pour les collectivités territoriales dont les recettes dépassent 100 millions d'euros ? En effet, la liberté d'organisation laissée aux présidents des chambres régionales et territoriales des comptes constitue une garantie d'indépendance des juridictions financières et permet de concentrer les contrôles sur les comptes présentant le plus de risques de dérapage. En outre, le renforcement des contrôles de gestion et la création du contrôle de l'annualité budgétaire pourraient représenter une charge supplémentaire non négligeable pour les CRC. De même, l'augmentation du nombre de justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière et la suppression de l'« ordre écrit » pour les fonctionnaires territoriaux conduiraient à à repenser le fonctionnement de cette cour qui rend moins de dix arrêts par an et dispose de moyens très limités. Or, comme l'a souligné Michel Delebarre dans son avis budgétaire sur les juridictions administratives et financières, le législateur a d'ores et déjà confié de nouvelles missions aux juridictions financières sans prévoir de moyens supplémentaires. Il conviendrait par conséquent de mieux évaluer l'effet concret de la proposition de loi sur la charge de travail des personnels de l'ensemble des CRC et de la Cour de discipline budgétaire et financière.

la présente proposition de loi : pour être sanctionnés, les élus locaux devaient avoir agi dans le cadre de leurs fonctions, avoir été informés de l'affaire et avoir donné l'instruction, quelle qu'en soit la forme, à un subordonné de commettre l'infraction. La commission des lois de l'Assemblée nationale avait étendu cette responsabilité financière aux ministres. Ce texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Les élus locaux doivent-ils être poursuivis devant la Cour de discipline budgétaire et financière pour des erreurs formelles dans l'application du droit budgétaire et comptable ? Ne conviendrait-il pas de redéfinir les infractions concernées ? Pourquoi ne pas étendre cette responsabilité aux ministres ? Enfin, il paraît difficile d'évaluer les conséquences de la suppression de l'« ordre écrit » pour les seuls fonctionnaires territoriaux.

Peut-on modifier le périmètre des justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière sans réformer, au préalable, le fonctionnement et le champ de compétence de cette juridiction ? Le projet de loi de 2009 prévoyait de supprimer cette juridiction, de transférer ses compétences à la Cour des comptes et de revoir l'ensemble des infractions sanctionnées. Plus récemment, M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, a souligné le manque de visibilité et d'efficacité de la Cour de discipline budgétaire et financière. Au terme d'un débat nourri, la commission des lois a jugé nécessaire d'approfondir sa réflexion sur la meilleure façon de renforcer la fiabilité des comptes des collectivités territoriales et de l'étendre à des problématiques plus larges, comme les moyens alloués aux juridictions financières et le rôle de la Cour de discipline budgétaire et financière. En conséquence, elle a décidé de déposer une motion tendant au renvoi à la commission de la proposition de loi et n'a pas adopté le texte. La parole est à M.

la proposition de loi présentée par votre collègue Vincent Delahaye. Ce texte, motivé par des situations locales observées après des changements d'exécutifs départementaux ou régionaux, comporte deux grands volets. Premièrement, un volet préventif vise à renforcer les contrôles. L'article 1 instaure une périodicité minimale pour le contrôle, par la chambre régionale des comptes, du respect du principe de l'annualité budgétaire par les collectivités territoriales les plus importantes et, ainsi, du dispositif de rattachement des charges Les modalités de ce contrôle seraient les suivantes un examen tous les deux ans, pour 112 collectivités dont les recettes dépassent 100 millions d'euros. En outre, un contrôle obligatoire des comptes et de la gestion s'appliquerait tous les six ans pour les collectivités les plus importantes. Deuxièmement, un volet répressif avec des sanctions nouvelles ou alourdies : ce texte propose en effet de rendre justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, la CDBF, les élus locaux au-delà de ce qui est déjà prévu aujourd'hui ; il renforce les sanctions applicables, le cas échéant, avec des peines d'inéligibilité ou pécuniaires, voire les deux, et crée comme corollaire un mécanisme de protection assurantielle des exécutifs locaux justiciables de la CDBF en cas de sanction pécuniaire. Les objectifs visés avec cette proposition de loi, c'est-à-dire la sincérité et la fiabilité des comptes locaux, sont totalement partagés par le Gouvernement. Je ne doute pas qu'ils le soient aussi par les membres de cette assemblée, car ils relèvent d'une exigence constitutionnelle. Je vais moi aussi citer l'article 47-2 de la Constitution Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Vous le savez, les comptes de l'État et des organismes de sécurité sociale sont d'ores et déjà certifiés. C'est aussi le cas, désormais, des comptes de la plupart des établissements publics nationaux, ainsi que des hôpitaux. Le secteur public local est moins avancé, c'est exact, mais une expérimentation de certification des comptes des collectivités locales a également été lancée. J'y reviendrai monsieur Delahaye, permet un échange de vues utile, et un point d'étape tout aussi utile sur ces chantiers très importants que sont la fiabilisation et la certification des comptes locaux. Cependant, je ne pense pas que les moyens que vous proposez pour y parvenir soient les plus adéquats. En effet, la systématisation du contrôle, par le juge financier, du rattachement des charges et des produits, qui est au coeur de votre proposition, présente, me semble-t-il, trois inconvénients. Elle nécessiterait tout d'abord des arbitrages délicats en termes de moyens alloués aux chambres régionales des comptes, les CRC. À ce stade, les conséquences potentielles en termes d'effectifs n'ont pas pu être expertisées finement avec la Cour Je vous rappelle que, en l'état, les contrôles des CRC sur les collectivités les plus importantes se font généralement tous les quatre ans. Ensuite, l'introduction de ce nouveau contrôle devrait aussi être articulée avec les dispositions actuelles relatives au contrôle budgétaire confié au préfet, et associant également les chambres régionales des comptes. Je rappelle que le contrôle budgétaire porte à ce stade sur cinq étapes du processus budgétaire : la date d'adoption du budget ; le respect de l'équilibre réel, ce qui renvoie à la question de la sincérité du budget ; la date d'adoption du compte administratif le déficit de celui-ci, et, enfin, l'omission ou l'insuffisance de crédits correspondant à des dépenses obligatoires. Par ailleurs, les exemples cités portent tous sur la question de l'annualité ou plus exactement du rattachement des charges et des produits à chaque exercice, prévu par les règles budgétaires et comptables. C'est vrai, cette thématique est importante, mais d'autres irrégularités, plus discrètes peut-être, peuvent aussi porter atteinte à la sincérité des comptes des collectivités territoriales. Il en est ainsi du défaut d'amortissement

C'est pourquoi, tout en partageant, je le répète, votre objectif, le Gouvernement privilégie une démarche différente, à la fois plus globale, c'est-à-dire visant à atteindre la qualité sur tout le champ comptable, et moins péremptoire, donc plus progressive et partenariale il ne suffit pas de généraliser les contrôles et de créer des sanctions ; il faut que les acteurs locaux s'approprient les bonnes pratiques. Des outils existent déjà, que le comptable public, et, au-delà, le réseau local de la direction générale des finances publiques, mettent à disposition des collectivités : restitution des contrôles comptables automatisés ; indicateurs de la qualité comptable locale. Ils donnent déjà une première tendance de la qualité des comptes. Mais, depuis 2011, pour agir plus en amont, la DGFiP travaille à fiabiliser les comptes locaux en relation étroite avec les associations d'élus. Il s'agit d'établir des guides ou référentiels de contrôle interne, qui permettent à l'ordonnateur de s'assurer que le budget comme la comptabilité sont tenus conformément aux règles en vigueur. Les thèmes de ces référentiels portent sur des sujets aussi divers et lourds de conséquences financières que les provisions pour risques et charges des collectivités, tout le cycle des recettes, l'évaluation du parc immobilier et les immobilisations financières. Ces travaux se déclinent aussi, sur le plan local, à travers la signature, avec le comptable public et la direction locale, de conventions de services comptables et financiers pour les collectivités les plus importantes ou, le cas échéant, d'engagements partenariaux pour les collectivités locales de taille plus modeste. Surtout, comme je l'ai déjà évoqué, le Gouvernement souhaite aller plus loin, ainsi que le prévoit la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, qui comporte une expérimentation de la certification des comptes sur 25 collectivités. Celles-ci ont été désignées en fin d'année dernière, parmi une cinquantaine de candidatures. Elles comprennent : 2 conseils régionaux, 6 conseils départementaux, 10 communes de taille variable et 7 EPCI, dont une métropole, situés tant en France métropolitaine que dans les territoires d'outre-mer. Pilotée par la Cour des comptes, mais associant naturellement dans sa mise en oeuvre le comptable public, la démarche de certification vise à porter une appréciation annuelle sur la qualité des comptes et repose sur la méthode suivante audit des processus à enjeux et analyse de la qualité des dispositifs de contrôle interne concourant à la fiabilité de l'information financière ; intervention d'auditeurs indépendants assujettis à des normes d'exercice professionnel reconnues, dont, le cas échéant, la dénonciation de faits délictueux « regard externe » d'un auditeur qui constitue un véritable levier de progression en matière de qualité comptable et conduit à une appréciation sur les états financiers annuels. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la proposition de loi dont vous débattez aujourd'hui a un objectif ambitieux, que le Gouvernement partage,

Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement donnera un avis favorable à la motion tendant au renvoi à la commission, ce qui permettra, je l'espère, de continuer à travailler les pistes contenues dans votre proposition,

il se trouve parfois, compte tenu de la durée de ces opérations, que c'est le successeur de l'auteur de l'erreur d'appréciation qui est ensuite amené à en assumer les conséquences. Bien entendu, ces dysfonctionnements méritent critique et suggèrent forcément des réflexions pour essayer d'y nous pouvons tous convenir que ce n'est pas uniquement à partir de ces éléments de circonstance, assortis en plus d'une certaine acrimonie politique, que nous pourrons inspirer la meilleure législation. Puisque le sujet a été évoqué, je veux donner ma propre lecture, partagée par mes amis, de ce qu'a été l'évolution de la législation dans ce domaine.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, qui ne peut partager le souci de sincérité et de transparence des comptes publics, en l'espèce des collectivités locales

Je suis convaincu, et même à peu près certain, que la très grande majorité des élus locaux, comme des fonctionnaires qui les assistent, est parfaitement respectueuse des règles comptables en vigueur pour ce qui est de la gestion locale. locale. Par conséquent, les errements constatés ne concernent que quelques situations bien connues. Je dois d'ailleurs souligner que, dans certains dossiers où des noms ont été en quelque sorte jetés en pâture à la vindicte populaire, les choses n'ont pas toujours été simples. Il ne suffit pas d'incriminer dans tous les cas les élus locaux, et eux seuls, ceux-ci ne déployant pas ou n'ayant pas déployé leur action dans un vase clos, sans interaction avec l'extérieur. Je pense, par exemple, aux collectivités locales victimes des emprunts structurés et de la montée en charge d'une dette libellée ou, à tout le moins, ajustée sur une devise étrangère s'étant quelque peu appréciée. Nous concevons fort bien le sens de l'article 1, qui tend à placer obligatoirement certaines collectivités, à compter d'un certain seuil de ressources, sous le contrôle attentif des chambres régionales des comptes, singulièrement en vue d'éviter la regrettable pratique de la cavalerie budgétaire. De même, nous pouvons concevoir de modifier les règles, voire le quantum des peines, si l'on peut dire, dès lors que la responsabilité des élus et des principaux fonctionnaires et cadres territoriaux les ayant assistés se trouve engagée quant à la situation de la collectivité ou de l'établissement public en difficulté. Nous sommes, en revanche, nettement plus circonspects, pour ne pas dire plus, devant le contenu de l'article 2, qui propose la mise en place, à terme, d'un dispositif d'assurance anti-sanction pécuniaire pour les élus locaux. On ne peut décemment, nous semble-t-il, appeler à la transparence et à l'éthique et imaginer dans le même temps un système qui, moyennant liquidation des primes versées par précaution, vous abriterait des foudres de la justice. L'élu « délinquant », si l'on peut dire, serait épargné au seul motif d'avoir été prévoyant ! Les errements qu'a pu connaître la gestion locale, notamment à Mennecy, dans le département de l'Essonne, dans les années 1990, à Yerres, dans les années 1980, à Bussy-Saint-Georges, apparemment également à Corbeil-Essonnes, sont parfaitement répréhensibles et ont été poursuivis comme tels. Il n'en demeure pas moins que tout cela pose aussi, et de nouveau, la question de la gestion locale, des marges de manoeuvre dont disposent les élus pour mener des politiques originales, et des moyens dont l'État dispose pour conseiller comme pour vérifier la qualité de la décision locale. Nous ne devons surtout jamais oublier, en dernière instance, que les habitants demeurent juges et parties. et parties. Par leurs impôts, la facturation des services rendus à la population, leur contribution directe et indirecte, ils financent les actions et les orientations politiques appliquées de leurs élus.

notamment parce que les plans d'apurement et de redressement comprennent toujours un volet fiscal. Songeons, pour donner quelques exemples, au cas des habitants d'Yerres, victimes des errements financiers d'un maire se piquant pourtant,

En 1995, un jeune maire fut élu à Yerres et mit en oeuvre un plan particulièrement sévère de redressement financier, qui fut confirmé, en quelque sorte, en 2001 Reconnaissons que les cures de redressement des comptes sont sévères et largement payées par la hausse des impôts locaux. Comment ne pas citer le cas de Saint-Cast-le-Guildo, cette petite ville balnéaire des Côtes-d'Armor où une équipe municipale, de sensibilité de gauche, mal conseillée, eut recours à un emprunt structuré conduisant à l'aggravation de l'endettement de la commune, avant qu'une alternance politique ne s'épuise à tenter de redresser la situation ? La responsabilité des élus n'a pas été formellement engagée, loin de là, dans cette affaire, mais la situation est telle que les électeurs ont, de nouveau, fait jouer l'alternance en 2014.

ce qui reste pour donner un cachet d'originalité à la gestion locale. Je suis convaincu que nos compatriotes attendent autre chose de leurs élus locaux que de se contenter de mener, en tout point du territoire, la même politique, en se préoccupant simplement de nettoyer les voies publiques, de les réparer et de les entretenir au besoin. Ils souhaitent, de manière légitime, que la politique menée dans leur ville ait un sens, une « couleur », qu'elle traduise des choix politiques originaux et clairs. clairs. Le moins que l'on puisse dire est que cela dépasse quelque peu la seule problématique soulevée par la présente proposition de loi. Au-delà de la transparence et de la sincérité souhaitées

mais il n'est la condition suffisante ni d'une saine gestion ni d'une gestion répondant aux besoins et aux attentes des populations. Le respect des règles comptables ne saurait, en dernière instance, être le seul mobile de la décision locale. Le renforcement des effectifs et de la qualité des agents de l'administration préfectorale est l'une des conditions de la résolution du problème. Avec des agents plus nombreux et mieux formés, cette administration sera mieux à même d'accomplir les missions qui lui sont confiées, notamment celle d'éclairer les élus locaux sur la pertinence de certains de leurs choix. De même, les services du Trésor disposent-ils des moyens matériels et humains pour faire face à la charge de gestion des comptes des collectivités locales de leur ressort ?

indique également qu'il est grand temps que la politique locale, comme la politique en général, reprenne quelque allure et que la démocratie participative, l'implication des citoyens et des citoyennes soient la base et la raison d'être de l'action locale. Quand les choix sont partagés, tout est plus clair

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous voudrez bien m'excuser de ne pas partager ce quasi-consensus sur la nécessité de renforcer les contrôles sur l'action des élus locaux. Appeler en renfort la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour justifier l'alourdissement de la tutelle sur des élus directement issus du suffrage populaire par des organismes sans autre légitimité démocratique que d'avoir été nommés par l'exécutif, il faut oser Mais, d'abandon de souveraineté au nom d'une Europe sans union en formalisme paralysant de la LOLF, de réformes comptables destinées à aligner la gestion publique sur la gestion privée en culte d'une illusoire transparence de papier, nous y sommes tellement habitués que nous trouvons naturel de faire certifier des comptes publics tenus à deux mains, l'une d'entre elles étant celle de fonctionnaires du ministère des finances, pour mieux sanctionner les ordonnateurs publics. Que de bruit pour rien ! », me dira-t-on. Cette proposition de loi appelle juste à un effort de vérité visant seulement à établir la situation financière exacte des collectivités annuellement et à sanctionner les ordonnateurs qui auraient manqué à leurs obligations, sans jugement sur les choix budgétaires des élus de la collectivité.

l'attention sur la conformité formelle des documents budgétaires aux règles comptables, ce que ne manquera pas de produire le spectacle médiatique qui entourera fatalement l'opération, c'est favoriser la confusion entre bonne gestion et régularité comptable, qui ne sont pas les mêmes choses. C'est imposer sans le dire une vision de la bonne gestion où l'endettement et les frais de personnel sont minimums, l'autofinancement maximum, quel qu'en puisse être l'intérêt réel pour les administrés, l'exposé des motifs. La qualité du service rendu, son coût, le poids réel de la fiscalité et son évolution, devenus secondaires, se perdront dans les commentaires annexes. Pouvoir dire que chaque habitant de telle commune ploie sous tant d'euros de dette et que les frais de personnels ont augmenté dans cette commune, voilà ce qui importera seul. L'impact réel de cette dette sur l'impôt de cette augmentation des frais de personnels sur le service rendu n'est pas la préoccupation des comptables, encore moins de ceux qu'ils nourrissent. On tient des chiffres comparables entre eux, donc susceptibles de faire les titres des gazettes : cela suffit. Qu'importe le reste ! J'irai plus loin

Je prendrai un exemple : l'introduction, pour les collectivités d'une certaine taille, de l'obligation d'amortir leurs investissements sur le modèle de la comptabilité privée, prise désormais comme modèle. Le caractère pervers de l'obligation d'amortir, c'est-à-dire de faire figurer en dépenses de fonctionnement une fraction des dépenses d'investissement, y compris les subventions d'équipement versées en toute liberté ce qui est pure stupidité, apparaît dès lors qu'elle conduit à interdire des dépenses utiles, simplement pour pouvoir garantir un niveau d'autofinancement purement décoratif. Ainsi, une collectivité présentant un excédent important de ses recettes réelles de fonctionnement sur ses dépenses réelles de fonctionnement peut se trouver contrainte, pour respecter le formalisme comptable, de réduire des dépenses de fonctionnement utiles. J'ai eu l'occasion de le constater avec effarement au temps où j'étais conseiller général

autres. Si l'on voulait vraiment répondre à l'attente de la société civile « en demande d'une éthique politique forte », plutôt que de compliquer un peu plus la vie d'élus croulant déjà sous les obligations, on pourrait peut-être

encore moins les procédures bureaucratiques. Elle retrouvera son dynamisme par ce qui fait sa force, à savoir le débat, la confrontation entre majorités et oppositions. Dotons donc les minorités des assemblées territoriales d'un statut leur permettant de jouer pleinement leur rôle, ce qui suppose un droit à l'information autre que celui dont elles disposent aujourd'hui. Or le fonctionnement des collectivités,

ces derniers étant trop souvent consternés par certaines attitudes déconsidérant l'ensemble des pratiques des élus.

il importe que les situations engendrant une certaine défiance puissent être répertoriées, identifiées et sanctionnées.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la France est à la traîne en matière de transparence des élus et de responsabilité en matière d'argent public

; elle est à la traîne de nombre de nos voisins européens, et la presse étrangère nous renvoie régulièrement l'image d'un pays à l'éthique aléatoire. Ce n'est pas sombrer dans le populisme que de reconnaître ce retard et de tenter de le combler. Cette proposition de loi s'inscrit dans ce mouvement justifié, en proposant de renforcer, d'une part, le contrôle de gestion des collectivités territoriales et, d'autre part, la responsabilité financière des élus locaux. Renforcer la périodicité du contrôle des plus grosses collectivités serait assurément bénéfique. Il faudrait simplement s'assurer que les chambres régionales et territoriales des comptes, les CRTC, aient les moyens de ce surcroît d'activité. Dans cet élan, nous pourrions d'ailleurs proposer que le Sénat, chambre des collectivités, soumette lui aussi sa gestion, à l'instar de l'Élysée, à un contrôle annuel de la Cour des comptes.

Nous devons assurer la transparence de notre institution, tout en respectant son indépendance. J'en reviens aux comptes des collectivités. Le texte vise également à créer un nouveau contrôle, fréquent et portant exclusivement sur l'annualité budgétaire.

et une telle focalisation se ferait nécessairement au détriment de contrôles plus exhaustifs. Vous avez expliqué le contraire, mon cher collègue, mais il faudrait dire comment on aurait le temps d'y procéder ! Ainsi, sur ce plan, il nous semble préférable de laisser aux CRTC la liberté de déterminer le périmètre de leurs contrôles. Ah ! Si nous devions attirer l'attention des CRTC sur un point, ce serait plutôt le contrôle des partenariats public-privé, qui comportent plus d'enjeux que les reports de charges. Les PPP ne sont toujours pas véritablement évalués par une instance indépendante, après que nos collègues Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli les ont qualifiés, dans un excellent rapport, d'« outils à haut risque » et de « bombes à retardement budgétaires ». La catastrophe des emprunts toxiques, qui a prospéré par manque de contrôle, devrait pourtant nous instruire. En ce qui concerne la responsabilité financière des élus locaux, on ne peut que partager la volonté de mettre fin à la différence de traitement entre les ordonnateurs, difficile à justifier. Ah ? En effet, les ordonnateurs qui appartiennent à la sphère politique - élus locaux et ministres -bénéficient d'une immunité partielle ou totale, alors que presque tous les autres ordonnateurs, notamment les fonctionnaires et membres de cabinet, sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière. Pour autant, la solution proposée, à savoir une extension de la compétence de la CDBF aux élus, nous semble incomplète. d'abord, la Cour n'aurait pas aujourd'hui les moyens d'assumer une telle extension. Sans doute faudrait-il d'ailleurs l'intégrer dans la structure juridictionnelle de la Cour des comptes et des CRTC, de manière à lui faire bénéficier des mêmes moyens et de la même déclinaison locale. Ensuite, par souci de cohérence et de justice, il paraît nécessaire de traiter en même temps le cas de tous les ordonnateurs, et en particulier des premiers d'entre eux, à savoir les membres du Gouvernement. Comment imaginer en Comment imaginer en effet que, pour une même infraction, le maire d'une petite commune soit passible d'inéligibilité, mais qu'un ministre ne puisse pas être poursuivi ? Telle serait pourtant la conséquence de cette proposition de loi. Par ailleurs, même si cette question ne relève plus du législateur national, on pourrait également s'interroger sur la situation de Mario Draghi, qui est devenu président de la BCE sans qu'aucune juridiction européenne ne soit saisie de son rôle, manifestement éminent, dans le maquillage des comptes de la Grèce par Goldman Sachs. Est-ce

n'est pas indépendant de ce qui se passe en France. Mais je laisse chacun à sa particularité locale et à sa volonté de ne pas dépasser le cadre national ... Enfin, sans doute faudrait-il remettre à plat l'ensemble des infractions et des peines imputables aux comptables comme aux ordonnateurs. Il serait utile de pouvoir mieux distinguer l'erreur bénigne de la faute sérieuse, et de leur associer des sanctions véritablement en adéquation. On pourrait aussi s'interroger sur la pertinence des sanctions pécuniaires, dont le montant dépend des sommes en jeu dans l'infraction. En conclusion, le groupe écologiste tient à saluer cette proposition de loi, qui pointe des lacunes avérées et relance l'intérêt pour la réforme des juridictions financières. Toutefois, chacun semble en convenir, la réflexion mérite d'être poursuivie, et surtout élargie.

C'est le résultat de situations constatées par nombre d'équipes majoritaires et d'exécutifs locaux, qui, passé la satisfaction et parfois l'euphorie de se voir confier l'initiative de préparer, d'examiner et de voter leur budget local, relèvent un certain nombre de manquements comptables ou budgétaires.

Ce type de dérives pose un vrai problème : certains exécutifs s'exonèrent de principes comptables fondamentaux, pratiques qui nuisent à la fiabilité et à la sincérité des comptes publics. Quand je pense que, en 2004, Ségolène Royal, fraîchement élue présidente de la région Poitou-Charentes, voulait créer d'elle-même un « observatoire des engagements » ! Celui-ci n'a n'a bien sûr jamais vu le jour. La même ne manquait jamais une occasion de proclamer, avec autant de gravité que de solennité, qu'« un euro dépensé est un euro utile » ! On sait maintenant qu'il fallait entendre : un euro engagé est un euro dissimulé

L'examen porte sur la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis en oeuvre dans l'utilisation des fonds publics et l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante.

examen annuel du respect de l'annualité budgétaire pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont les recettes sont supérieures à 200 millions d'euros par an, qui s'ajoutera à la vérification de leurs comptes tous les six ans. Pour les collectivités territoriales dont les recettes sont supérieures à 100 millions d'euros par an, mais inférieures à 200 millions d'euros par an, un contrôle annuel limité serait effectué tous les deux ans. La transmission obligatoire des irrégularités constatées par la CRC à la Cour de discipline

aussi parfois, il faut le dire, que l'erreur constatée ne soit pas commise sciemment dans le but de dissimuler la réalité des comptes de la collectivité locale. C'est pourquoi la motion de renvoi en commission semble opportune.

et l'expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales. C'est pourquoi la commission appelle, à juste titre, à choisir entre ces deux procédures pour éviter un « empilement malvenu des dispositifs de fiabilisation des comptes locaux. Il convient donc bien, me semble-t-il, d'attendre le bilan d'étape de l'expérimentation de certification des comptes, dont la publication est prévue l'année prochaine, afin,, de pouvoir évaluer au mieux l'intérêt de chacune de ces procédures.

je remercie nos collègues Vincent Delahaye et Catherine Di Folco pour le travail effectué sur cette proposition de loi visant à assurer la sincérité et la fiabilité des comptes des collectivités territoriales. L'article 47-2 de la Constitution dispose que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. En réalité, il est très difficile de répondre à cette exigence légitime. Les élus et les agents territoriaux, mais aussi les comptables publics, s'impliquent constamment et avec détermination en cette matière, mais la fiabilité des comptes locaux reste perfectible. Il est vrai que des exemples concrets viennent alimenter la thèse d'un besoin de perfectionner la fiabilité des comptes des collectivités. Je pense notamment aux trois cas de « doutes

Des retards de paiement auraient été pratiqués de manière systématique et auraient permis de reporter d'une année sur l'autre jusqu'à 10 % des dépenses de fonctionnement. Comment, au regard de ces trois exemples, peut-on ne pas douter de la sincérité des comptes ? Il nous faut, nous, élus, être plus que jamais responsables ! Ce texte prévoit un volet préventif, à savoir le renforcement des contrôles non juridictionnels des chambres régionales et territoriales des comptes, et un volet répressif, à savoir l'élargissement des compétences de la Cour de discipline budgétaire et financière. Le texte prévoit également une saisine automatique du ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière lorsque les chambres régionales et territoriales des comptes constatent, à l'occasion d'un contrôle de gestion ou d'un contrôle de l'annualité budgétaire, une infraction sanctionnée par cette juridiction. Les chambres régionales et territoriales auraient l'obligation de contrôler, au moins tous les six ans, la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dont les recettes annuelles dépassent régulièrement 200 millions d'euros, soit près de 200 collectivités territoriales et établissements publics. Les chambres régionales et territoriales des comptes seraient également chargées d'examiner le respect du rattachement des charges à l'exercice budgétaire en cours, conformément au principe de l'annualité budgétaire, et cela tous les ans pour les collectivités territoriales dont les recettes dépassent régulièrement 200 millions d'euros.

Il conviendrait de mieux traiter l'impact concret d'une adoption de la proposition de loi sur la charge de travail du personnel de l'ensemble des chambres régionales et territoriales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière.

Un autre point de ce texte peut susciter des interrogations : le rôle et les compétences de la Cour de discipline budgétaire et financière. On peut en outre s'interroger sur la mise en oeuvre de la responsabilité des élus locaux devant cette cour. Par exemple, une simple erreur dans l'application des règles budgétaires et comptables, lesquelles sont par ailleurs de plus en plus complexes, ne me semble pas justifier l'engagement de leur responsabilité personnelle. La peine de cinq ans d'inéligibilité me paraît elle aussi disproportionnée.

D'ailleurs, cette proposition de loi revient sur un principe de base de la décentralisation : en l'état actuel du droit, le contrôle s'exerce. En revanche, réformer le fonctionnement et le champ de compétences de la Cour de discipline budgétaire La rapporteur nous l'a confirmé, à la suite des auditions qu'elle a pu mener : cette juridiction manque de visibilité et d'efficacité. Je rappelle qu'en 2009 un projet de loi inspiré par Philippe Séguin, alors Premier président de la Cour des comptes, prévoyait la suppression de la CDBF et le transfert de ses compétences à la Cour. Un point

L'examen de la gestion est un contrôle mal calibré par rapport à son objectif. Il est censé constituer un instrument d'aide à la gestion pour les collectivités. Or les élus ont de plus en plus de mal à percevoir sa valeur ajoutée par rapport à l'expertise dont ils disposent au sein de leur administration. L'exercice est pourtant très lourd, pour les élus comme pour les chambres. Aussi la procédure telle qu'elle est conçue aujourd'hui est-elle inadaptée. Elle peut durer jusqu'à trois, voire quatre années, avec plusieurs conséquences regrettables : la mobilisation des personnels de la collectivité et de la chambre pendant une telle durée, le risque accru d'un changement d'interlocuteurs en cours de procédure, un fort décalage temporel entre la période examinée et la remise des observations. En tout état de cause, ce sujet devra être lui aussi approfondi afin d'alléger la procédure ou du moins de la clarifier. On constate en effet dans de nombreuses communes que ces contrôles se font de manière assez aléatoire, et surtout mobilisent une énergie considérable des agents des collectivités. À mon sens, il est nécessaire de redéfinir les priorités de contrôle des chambres régionales et territoriales des comptes, afin qu'elles soient plus homogènes, et de s'assurer que les collectivités dont les comptes sont situés en dessous du seuil actuel des « comptes significatifs » ne soient pas exclues d'un tel contrôle de manière systématique. Enfin, et pour conclure, il est évidemment préférable d'attendre le rapport relatif à l'expérimentation de certification des comptes des collectivités territoriales prévu par la loi NOTRe, qui doit être rendu public en 2018. L'esprit de cette proposition de loi est tout à fait honorable, mais il est nécessaire à la fois d'être patient, notamment au regard de la loi NOTRe, et d'approfondir un sujet qui a suscité de nombreuses interrogations, tant en commission qu'aujourd'hui, dans l'hémicycle. La parole

une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». Nos collègues soulignent en particulier plusieurs cas dans lesquels des « doutes sérieux » ont été exprimés sur la sincérité des comptes présentés par les collectivités territoriales. Ils souhaitent organiser un cadre légal afin d'éviter que ce type de situation ne se reproduise à l'avenir.

Ne serait-il donc pas incohérent et précipité de prévoir d'ores et déjà le contrôle de l'annualité budgétaire, avant même que les leçons à tirer de cette expérimentation soient connues ?

D'un point de vue institutionnel, il ne serait pas anodin de soumettre les élus locaux à un tel contrôle et de faire peser une telle responsabilité sur leurs épaules. leurs épaules. Il y a tout juste trois mois, le Conseil constitutionnel a jugé conforme le régime d'exemption applicable aux élus locaux à l'égard de la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le bilan du quinquennat est très lourd et en partie destructeur parce qu'imposé sans cadre négocié pour traiter des finances de nos collectivités territoriales : ces dernières ont vu le montant de leurs dotations

Nos élus, qui exercent une fonction exigeante, se trouvent donc pour beaucoup confrontés à de graves difficultés financières dans les collectivités dont ils ont la responsabilité. Bien sûr, il n'est en aucun cas

Dans son rapport annuel de 2015, la Cour de comptes relevait déjà des imperfections et des insuffisances dans la présentation des comptes de certaines collectivités territoriales, qui manquaient de fiabilité et de clarté. Elle remarquait également, « au-delà des difficultés liées à l'équilibre budgétaire, une méconnaissance, voire une incompréhension, des règles applicables ». N'y aurait-il pas là une source de réflexions pour la commission des lois ?

satisfaire une exigence de transparence à l'égard de nos concitoyens, en assurant la présentation de comptes fiables, clairs et sincères ; à cette fin, prévoir, pour les élus et leur personnel, des outils faciles d'utilisation et d'accès. C'est un travail minutieux que la commission des lois est invitée à fournir pour atteindre cet objectif. Ces outils devraient en effet être adaptés à tous les profils et tailles de collectivités. Le tome II du rapport sur l'évolution des finances locales à l'horizon 2017, présenté par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation en juillet 2015, ne démontrait pas autre chose les consultations des élus locaux révélaient que ces derniers souhaitaient un étalement des baisses de dotations dans le temps et une simplification de la fiscalité locale. La réforme de la dotation globale de fonctionnement, dont il a été si longtemps question, a été reportée par le Gouvernement.